bien vouloir excuser l'absence du président du Sénat, qui assiste aujourd'hui au Congrès des maires de France. On peut applaudir tous nos collègues maires. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer, au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect des uns et des autres et celui du temps de parole.

Malgré l'instauration d'un couvre-feu, l'île de la Réunion reste encore aujourd'hui le théâtre d'une flambée de violences urbaines. De nombreux services publics, entreprises et commerces sont bloqués ou inaccessibles. J'ai entendu le message du Président de la République hier soir, mais la répression ne doit, en aucune manière, être la seule réponse apportée par le Gouvernement

Des mesures fortes doivent être prises immédiatement. Le gel de la taxe sur le carburant décidé par la région de la Réunion est une première réponse, mais l'État doit aussi agir et la compléter.

Il faut aussi soutenir les entreprises et revoir les seuils retenus pour le calcul des exonérations prévues dans le cadre de la réforme des aides économiques. Ces mesures sont non pas des avantages indus, mais une nécessité ! Elles sont le reflet des sujétions et des spécificités de l'outre-mer.

La Réunion, vous l'avez dit, connaît depuis samedi soir un climat de tension extrême. Des actes graves ont été commis contre des dépositaires de l'ordre public. Nous estimons tous ici que c'est intolérable. En matière de sécurité, nous apportons une réponse juste et mesurée. Près de 110 casseurs ont été interpellés. Certains ont été lourdement condamnés en comparution immédiate. Je le redis ici, des actes intolérables ont été commis et ils devront être punis.

Un an après, les chiffres des neuf premiers mois de l'année viennent de tomber. Tous les experts- je dis bien : tous les experts ! -sont d'accord pour dire que la construction neuve va connaître une récession grave dans les zones urbaines et très grave dans les campagnes et dans les villes moyennes. La situation est si grave que le P-DG de Nexity a publié une lettre ouverte au Président de la République dans les journaux et que le président de la Fédération du bâtiment vient de déclarer qu'on allait tout droit vers une crise. Il annonce la perte probable de 200 000 emplois dans le bâtiment à l'horizon de 2020.

Pour faire baisser le prix du logement et relancer la demande, allez-vous inverser vos mesures fiscales afin de ne pas nous faire perdre, comme en 2014, un demi-point de croissance et de ne pas nous conduire tout droit dans le mur l'année prochaine et l'année suivante ?

s'associe ma collègue Viviane Malet, s'adresse à deux ministres ici présents. Si un début de réponse a été apporté aux événements quasi insurrectionnels de La Réunion, quelles réponses sont apportées à la souffrance exprimée par les « gilets jaunes » ? Comment en est-on arrivé là, et à qui la faute ?

saigne ... La mise en oeuvre de vos réformes pâtit d'un gros défaut de synchronisation et d'un manque de dialogue évident avec les élus de France, qui vous lancent pourtant régulièrement sur ces travées un avis de tempête.

Samedi 17 novembre, nombre de Réunionnais ont exprimé leur mécontentement à l'égard, entre autres, de la hausse des prix du carburant par une forte mobilisation. Ce mécontentement, pacifique au départ, a rapidement dégénéré en une flambée de violences qui paralyse l'île. Tous les établissements scolaires, des crèches à l'université, ainsi que les administrations locales sont fermées. La quasi-totalité des événements culturels et sportifs sont annulés. Un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes jusqu'à vendredi au moins. Il sera interdit d'y circuler entre vingt et une heures et six heures du matin. Si nous déplorons et condamnons évidemment les actes de violence et les pillages commis en marge des manifestations pacifiques, nous devons néanmoins entendre et écouter les messages envoyés par la population. La paralysie que nous connaissons est encore plus grave qu'en métropole. Comme vous l'avez justement dit, madame la ministre, La Réunion est le département le plus inégalitaire. À ma demande, vous avez accepté une rencontre avec les élus réunionnais lundi soir au Sénat. Cet échange constructif n'a pas pu se prolonger sur le terrain. En effet, contrairement à vous, qui dialoguez avec nous, le préfet a refusé d'entamer un dialogue avec les représentants du mouvement, alors qu'il les avait invités. Ce comportement du représentant de l'État est vécu comme une humiliation par les Réunionnais. Au nom de tous les parlementaires et élus locaux réunionnais, je vous invite à venir à La Réunion le plus rapidement possible, car nous savons que le dialogue est possible avec vous. J'en viens à ma question. Madame la ministre, que compte faire le Gouvernement pour rétablir les conditions d'un véritable dialogue entre l'État et la population réunionnaise, afin que la situation s'apaise et que des solutions pérennes puissent être trouvées ? La parole

des revendications des « gilets jaunes ». Sur le premier point, je veux ici de nouveau dire tout mon soutien aux forces de l'ordre, qui travaillent chaque nuit à rétablir la sécurité

Mesdames, messieurs les ministres, je peux comprendre que vous vous lassiez du jaune ces jours-ci ; aussi, je vais vous proposer de l'orange ! Chacun salue évidemment le développement du groupe Orange à l'international,

Comment expliquer que des fils tombés restent à terre plusieurs mois ? Ces défaillances ont des conséquences sur le quotidien des Français et sur leur capacité à joindre les services d'urgence dans des zones où, précisément, la couverture mobile est encore défaillante. Nous connaissons les plans en cours, monsieur le ministre, mais nous vous demandons solennellement, à double titre, en tant qu'actionnaire, d'une part, et en tant que gardien d'une mission de service public, d'autre part,

J'ai donc demandé à Orange de nous proposer un plan d'action. Mes services recevront Orange dans quelques jours pour en vérifier la viabilité. De deux choses l'une soit Orange est capable de remplir ses obligations, telles qu'elles ont été fixées par arrêté et telles qu'elles sont contrôlées par l'ARCEP, en déployant toutes les équipes nécessaires sur le terrain- je rends hommage au passage aux équipes d'Orange qui se démènent pour faire le maximum

j'ai besoin de vous parce que le pays ne se redressera pas avec quelques décisions, quelques lois, quelques règlements ou l'action de quelques-uns. Il ne réussira que parce que, partout sur le territoire, il y a les engagés et les convaincus que vous êtes. « Rien ne sera possible sans cette relation de confiance et de responsabilité. Ainsi parlait Emmanuel Macron devant les maires de France il y a juste une année. C'est beau comme l'Antique Si ce n'est que la défiance s'est depuis installée entre le pouvoir et les élus, défiance qu'un geste hautement symbolique permettrait de dissiper, au moins partiellement : inscrire dans la loi, enfin, un statut de l'élu territorial à la hauteur des attentes et, surtout, des besoins. Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à faire ce geste ?

Monsieur le ministre de l'impossible, les constats ne remplacent pas les actes et les promesses sont toujours à crédit

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus d'élus de nos communes rurales, maires, mais aussi conseillers municipaux, traversent une véritable crise des vocations, au point de démissionner de plus en plus en cours de mandat. On parle d'un « blues » des maires. Loin d'être un simple vague à l'âme, il s'agit d'une réelle lassitude. En tant que sénatrice et élue des territoires, je ne peux qu'être alarmée face à une telle désaffection, qui fragilise nos départements et risque de laisser nos concitoyens les plus isolés, pour lesquels le maire est souvent le seul référent politique et social, dans un grand désarroi. Baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation, organisation territoriale de plus en plus complexe, poids des intercommunalités : les raisons de quitter la fonction de maire ne manquent pas et s'accumulent. Nos élus doivent gérer un budget de plus en plus contraint et des politiques publiques qui manquent souvent de lisibilité. On leur demande toujours davantage ; on continue de les solliciter localement sur certains sujets, tout en leur ôtant l'autonomie et les moyens financiers pour ce faire. Or les maires de nos petites communes accomplissent un travail remarquable et très souvent de façon bénévole. Le manque de considération de l'État à leur égard nourrit légitimement ce sentiment de découragement et d'abandon. Le Sénat a présenté plusieurs rapports assortis de recommandations afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, ou encore pour conforter et revitaliser le rôle des communes, cellules de base de la démocratie. Monsieur le ministre, comment comptez-vous redonner aux maires la place qui leur revient de trait d'union entre les territoires et l'État et, surtout, les moyens de répondre aux attentes de nos concitoyens ?

Oserais-je vous dire qu'ayant été maire de 2008 à 2018 et conseiller municipal à partir de 1995 j'ai l'impression que ce n'est pas le bilan de ce gouvernement que vous dressez

prochain, sur le sens des mesures que nous prenons afin de faciliter la transition des territoires. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui un certain nombre de transitions pour la reconquête industrielle. Il n'y a pas d'avenir dans les territoires ni d'espoir pour les élus sans reconquête industrielle. C'est l'ensemble de ces leviers qu'il nous faut activer, et je suis sûr que le Sénat nous encouragera

Monsieur le ministre, Porte de Versailles, les maires sont moroses, dénonçant une absence de visibilité sur le plan de la fiscalité locale et encore abasourdis par le traitement que leur a réservé le prélèvement à la source. Absence de visibilité, car, si le projet de loi de finances garantit techniquement l'enveloppe globale de leurs dotations, ils décèlent des variations incontrôlées ; c'est tout un système qui prend l'eau avec l'inconnue des ressources de remplacement de la taxe d'habitation et le renvoi à une loi de finances exceptionnelle à venir en 2019, alors qu'ils remarquent les réparations d'urgence de la dotation d'intercommunalité et assistent au jeu de bonneteau entre les ressources de la métropole du Grand Paris et les établissements publics la composant. Première question, monsieur le ministre, afin de faire cesser cette incertitude, pouvez-vous leur dire si le PLF 2019 attendu se limitera au simple ajustement du remplacement de la taxe d'habitation ou s'il engagera,, les bases d'une véritable réforme d'ensemble ? Par ailleurs, les maires restent très attachés au caractère spécifique de leur mission auprès de leurs administrés. Jusqu'alors, à ce titre, ils bénéficiaient d'un régime d'exonération de leurs indemnités et compensant leurs frais engagés, jusqu'à l'équivalent d'un maire de 2 000 habitants et plus. Le prélèvement à la source ramène ce seuil au niveau du maire de 500 habitants et les assimile à des salariés purs et simples. Allez-vous les aider en favorisant notre demande très concrète de leur rendre justice, en rétablissant ce statut particulier auquel ils demeurent très attachés

le système établi voilà plus de cinquante ans ne pourra supporter le cumul des suppressions de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation. Vous êtes là pour gouverner et vos propositions tardent trop à cet égard. Vous ne semblez pas appréhender totalement le problème des indemnités et du statut de l'élu, mais je vous accorde le bénéfice du doute et vous en recommande une seconde lecture plus attentive, en attendant nos propositions.

Des sujets majeurs sont absents : la révision de certains périmètres de groupements hospitaliers de territoires, la réorganisation des organismes d'État, le soutien des carrières hospitalières. Si votre plan favorise la coordination des différents acteurs, il n'en reste pas moins que les infirmiers s'en sentent exclus. La mise en place des assistants médicaux pose question. La désespérance et l'épuisement règnent dans la majorité des hôpitaux publics. Ainsi, 78 % des présidents de centres hospitaliers estiment que leur établissement sera en déficit en 2018 43 % annoncent un déficit supérieur à 3 %. Dans mon département, le Lot-et-Garonne, les trois hôpitaux sont en déficit. Faire plus avec moins, c'est insoutenable ! C'est une politique qui touche l'hôpital, comme nos collectivités. Une pause doit donc être opérée sur les économies demandées. Il faut mettre fin aux fermetures de lits. Nous attendons la mise en oeuvre de votre plan et nous espérons que les effets seront bénéfiques. Pour le moment, les difficultés liées à l'attractivité médicale touchent 87 % des établissements ; cette situation conduira inéluctablement à une rupture irréversible de notre offre de soins. Madame la secrétaire d'État, quel avenir pour les infirmières et les infirmiers ? L'hôpital public peut-il compter sur une accélération des mesures et une anticipation des situations ? Naviguer à vue, comme le montre l'examen de la proposition de loi visant à sécuriser l'exercice des praticiens diplômés hors Union européenne est plus que préoccupant. Vous le savez, sans ces praticiens, les petits hôpitaux de nos départements ruraux fermeront les uns après les autres. La parole

non, les infirmières et les infirmiers ne sont pas oubliés, ils sont bien partie intégrante du plan « Ma santé 2022 ». Oui, il existe un malaise chez les professionnels de santé, notamment les infirmiers, qui n'est malheureusement pas récent, qu'il ne faut pas ignorer et que nous n'ignorons pas. En réalité, ce malaise est le symptôme d'un système de santé qui n'est plus adapté aux besoins de santé, qui n'est plus lié aux défis du XXIsiècle et qu'il faut profondément transformer. Cette transformation en profondeur est au coeur du projet porté par le Gouvernement, qui est non pas une liste de mesures catégorielles, mais une vision à long terme de notre système de santé, où chacun a nécessairement sa place.

nous souhaitons mettre fin aux logiques de cloisonnement des professionnels de santé. Nous développons de nouvelles compétences pour les infirmiers. La reconnaissance des infirmiers en pratique avancée est une évolution majeure pour notre système de santé, que nous avons mise en place à leur demande. Dix formations en centres universitaires seront également mises en place, dès la rentrée 2018, à leur demande. Nous élargissons leurs missions de prévention, notamment en matière de vaccination, avec l'élargissement des compétences à la primo-vaccination contre la grippe. Les représentants des infirmiers doivent retrouver le chemin des accords conventionnels avec la reprise des négociations conventionnelles,

nous sommes dans une semaine importante pour les élus de nos territoires, la semaine du Congrès des maires à Paris. Cette semaine est importante à double titre : c'est le moment où les maires se rencontrent, échangent, participent à des colloques, sous l'égide de l'Association des maires de France. En parallèle, c'est un temps où le Gouvernement écoute et entend leurs préoccupations, éclaircit des orientations et tisse la relation de confiance indispensable entre la représentation locale et la représentation nationale. Je sais que vous attachez une grande importance à la relation avec ces élus et les différentes associations qui les représentent. Mme la ministre Jacqueline Gourault est d'ailleurs récemment venue à la rencontre des élus drômois lors du congrès des maires Les maires l'ont interrogée, écoutée et ils ont apprécié ses jugements. Depuis quelques jours en effet, les Français reçoivent leur taxe d'habitation. Pour une part significative d'entre eux, ils voient cet impôt baisser sur leur avis d'imposition dès cette année et ainsi augmenter leur pouvoir d'achat. d'achat. C'était une promesse de campagne, elle est tenue. Dans le même temps, vous le savez, les maires s'interrogent sur la façon dont cette ressource communale va être compensée par l'État, non seulement à court terme, mais aussi pour les années à venir. Les maires d'aujourd'hui, comme ceux qui seront élus en 2020, ont besoin de lisibilité sur l'évolution de leurs ressources pour programmer leurs projets. À l'heure où nous débattons du projet de loi de finances pour 2019, pouvez-vous nous indiquer comment le Gouvernement envisage de compenser et de préserver des ressources dynamiques dans la durée ?

Gouvernement. Vous avez raison, et vous l'avez bien décrit, le Congrès des maires est un moment important pour nos élus : c'est un moment de dialogue, un moment pour faire le point sur la situation de nos collectivités locales, tout particulièrement des mairies, un moment aussi pour se projeter et regarder l'avenir, l'avenir territorial et fiscal, avec les finances des collectivités locales. Le Président de la République l'a rappelé dans un courrier adressé à l'ensemble des maires de France et dans un échange qu'il a eu hier avec près de 2 000 maires au Palais de l'Élysée. Un « échange » ? Le Premier ministre est en train de faire un discours où il exposera la politique du Gouvernement. Vous m'interrogez sur la suppression de la taxe d'habitation.

Ma question s'adresse à Mme la ministre des outre-mer. J'aimerais m'associer aux questions posées par nos collègues de l'île de la Réunion. Il faut effectivement rester attentif à la situation explosive que vit l'île, qui est, au moment où nous parlons, sous le régime d'un couvre-feu. J'exhorte le Gouvernement, au-delà de la nécessité du maintien de l'ordre, à ne pas prioriser la seule réponse répressive et donc à engager un dialogue. J'ai entendu notre collègue Michel Dennemont dire que le représentant de l'État n'a pas voulu recevoir les manifestants ou les collectifs. Connaissant la conflictualité sociale de nos îles, il faut absolument prioriser le dialogue. C'est un voeu que nous émettons, le groupe socialiste et

est ma réponse et celle que pourrait vous apporter Mme Annick Girardin. Ce sont, à périmètre constant, les crédits supplémentaires dont vont bénéficier tous les territoires d'outre-mer pour l'année 2019, avec une volonté du Gouvernement de réorienter ces crédits d'abord vers l'activité économique et les entreprises, pour créer de l'emploi et répondre au chômage de masse, dont vous conviendrez qu'il est aujourd'hui la première faiblesse et le premier drame des territoires d'outre-mer. Par ailleurs, les territoires d'outre-mer bénéficieront, comme tous les autres territoires français, de la suppression de la taxe d'habitation, des mesures qui sont prises pour soutenir l'emploi et ceux qui travaillent.

Eh bien, moi, je voudrais pointer une contradiction française, qui est celle de vouloir à la fois réduire les impôts et demander toujours plus de dépenses publiques Cette contradiction ne peut être résolue qu'avec la politique dans laquelle nous sommes engagés avec le Président de la République et le Premier ministre. Si nous voulons baisser les impôts, il faut soutenir la croissance et réduire la dépense publique. Soutenir la croissance, c'est ce que nous faisons avec une fiscalité favorable aux entreprises, à l'investissement, à l'innovation, qui nous permet de baisser le chômage de 0,5 point depuis un an, et c'est soutenir le travail en le rémunérant mieux : tous les salariés français ont vu au 1 novembre que leur salaire net avait augmenté. Et réduire la dépense publique, c'est avoir le courage de voter des décisions difficiles sur les emplois aidés, les chambres de commerce et d'industrie, l'audiovisuel public, pour parvenir à réduire la dépense, diminuer la dette et poursuivre la baisse des impôts. Nous tiendrons le cap de un point d'imposition en moins et de prélèvements obligatoires en moins pour l'ensemble des Français. Dans ces temps agités,

la création d'emplois et en tenant le cap de la réduction de la dépense et de la dette que nous redresserons la France, pas avec des mesures de court terme, pas avec plus de dépenses et plus de dettes ! La parole est

je l'avoue ! Le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à octroyer, après analyse, 4,5 milliards d'euros aux outre-mer pour corriger le mal-développement,

avec la culture qui est celle du Sénat, à avoir le sens du dialogue, à trouver les compromis raisonnables que nous ne manquerons pas de vous proposer et qui, je l'espère, auront l'agrément de tous les groupes de cette assemblée.

Monsieur le ministre, l'an I du nouveau monde a vu l'avènement d'une de vos oeuvres inachevées : la Conférence nationale des territoires, qui devait, selon le Président de la République, bâtir un pacte de confiance. Mais, comme il arrive parfois, hélas, dans une discussion, les élus ne sont pas venus vous dire ce que vous vouliez entendre. En revanche, eux ont entendu vos promesses rassurantes, démenties avec une célérité qui, je dois le dire, force le respect. Las de ne pas être écoutés, les élus ont lancé un appel, celui de Marseille, resté quasiment sans réponse, si ce n'est un catalogue de bonnes intentions. Pourtant, ils avaient pris au sérieux le Président de la République quand, sûrement dans un moment d'égarement, celui-ci leur déclarait, il y a un an, au Congrès des maires

lorsqu'on sait que la majorité d'entre eux ne souhaitent plus s'investir après 2020. Le candidat En Marche rêvait de changer le personnel politique, le Président Macron pourrait, malheureusement, être comblé ! Ma question est donc simple : alors que le dialogue est au point mort sans que de réelles avancées aient vu le jour, qu'envisagez-vous concrètement pour l'avenir de nos communes ?

Vous reconnaîtrez, monsieur le sénateur, que l'exercice auquel s'est prêté le Président de la République hier était non pas un dialogue artificiel,

et une vraie écoute, et non pas simplement un discours qu'il faut faire parfois devant les associations d'élus, mais qui, reconnaissons-le, ne prête pas beaucoup au dialogue. Vous m'interrogez par ailleurs sur la Conférence nationale des territoires.

un format complet présidé par le Premier ministre, un format restreint ou bureau, sous la présidence de la ministre de la cohésion des territoires, qui réunira les présidents des deux délégations parlementaires et un représentant de chaque association d'élus. Paroles, paroles ... Le Gouvernement souhaite que chaque association d'élus y soit représentée. Enfin, des groupes thématiques y seront

Ma question était destinée à M. le Premier ministre. Que de chemin parcouru depuis 2017 ! J'entends encore vos slogans de campagne : « Il faut en finir avec le " vieux monde " » ; « il faut remettre les Français au coeur de la vie politique les Français attendent que les pratiques de leurs responsables politiques deviennent plus représentatives, plus responsables et plus efficaces » ... Monsieur le Premier ministre, avez-vous objectivement l'impression d'avoir atteint ces objectifs ? J'entends les retraités, les automobilistes avec les 80 kilomètres par heure, certains de vos députés, les conseillers départementaux, et bien d'autres. Tous déçus J'entends ces « gilets jaunes », ces familles qui n'ont jamais manifesté, mais qui ne supportent plus l'augmentation des carburants et des taxes, ces familles qui travaillent mais sont à découvert dès le 20 du mois. J'entends aussi ces maires, qui ont perdu leur liberté d'agir et dont les budgets sont en baisse, mais qui restent responsables de tout, y compris des catastrophes, ces maires écoeurés qui ne veulent pas renouveler leur mandat en 2020. Vous entendez, monsieur le Premier ministre, mais vous n'écoutez pas ! De plus en plus, nous avons l'impression d'être tous ensemble dans un avion. Le Président de la République et vous-même, monsieur le Premier ministre, enfermés dans le cockpit ; les Français, tous passagers ! Aux commandes, vous luttez pour ne pas perdre de l'altitude. Mais rien n'y fait la croissance est en berne, le chômage reste au même niveau, la balance du commerce extérieur est toujours négative, les dépenses de l'État augmentent, le sentiment d'insécurité persiste. La porte est close ; vous ne répondez plus aux passagers, qui s'inquiètent ! Vous envoyez pourtant par moment vos chefs de cabine, comme Mme le ministre de la cohésion des territoires, pour nous dire que tout va bien, ou le ministre de l'intérieur, pour vérifier que nos ceintures sont bien attachées et que personne ne bouge. Même votre ancien ministre de l'intérieur l'a compris et a pris son parachute ! Quand allez-vous comprendre que vous n'y arriverez pas seuls ?

Il n'est pas acceptable d'insulter, d'intimider ou de menacer des élus locaux ou des élus de la Nation. Il n'est pas acceptable de voir fleurir sur des réseaux sociaux des appels à la haine ou à la destruction.

Merci

nous entamons aujourd'hui l'examen du deuxième projet de loi de finances du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous l'examinons dans des conditions particulières. La société française connaît des tensions exacerbées, latentes depuis de nombreuses années, mais qui s'expriment aujourd'hui concrètement, jusque dans la rue. Face à ces tensions, nous devons examiner la situation budgétaire du pays et les solutions à apporter, sans excès, sans caricature, avec responsabilité et modération. Il importe de regarder les choses de façon pragmatique. C'est la raison d'être du groupe Les Indépendants. En somme, je vous propose de regarder les choses telles qu'elles sont et de débattre sur des faits et des valeurs. Et sur des chiffres aussi ! Quelles sont les valeurs du groupe Les Indépendants ? La justice sociale, la responsabilité budgétaire et une efficacité économique qui doit être mise au service de tous. J'ajouterai que nous sommes en faveur d'un développement durable sur le long terme, pragmatique et réaliste, adapté au quotidien de tous les Français.

Oui, il faut changer de modèle de société. Oui, il faut favoriser la transition énergétique. Oui, il faut tenir bon sur les ambitions climatiques qui sont les nôtres- elles sont nécessaires et légitimes mais il faut le faire avec pragmatisme et pédagogie. Il faut nous assurer que personne n'est laissé au bord du chemin de l'écologie, un chemin que nous soutenons et que nous jugeons nécessaire. Nous aurons donc à coeur, sur cette question, de proposer des alternatives crédibles à des hausses de taxe indiscriminées et parfois incohérentes. Il faut sortir de la logique punitive perçue par nos concitoyens ou nos PME. Notre responsabilité est de démontrer que la transition écologique est une chance pour chacune et chacun des Français.

Cette exigence doit dès à présent être intégrée au fonctionnement même de l'État. Nous demanderons ainsi au Gouvernement d'introduire le respect des « objectifs du développement durable » de l'ONU dans le processus budgétaire, pour éclairer l'orientation des grandes politiques publiques. Ce projet de loi de finances est également le véhicule de réformes majeures pour nos entreprises. Je pense bien sûr à la fiscalité des brevets et de l'innovation, pour l'adapter aux exigences de l'OCDE.

veiller à la stabilité et à la sécurité juridique indispensables au développement des entreprises. Ensuite, les législateurs que nous sommes ne doivent pas avoir la main trop lourde dans la transposition d'exigences internationales. Nous devons veiller à préserver la compétitivité de nos entreprises et de nos centres de recherche en Europe et dans le monde. Enfin, il faut absolument respecter la spécificité des PME et des entreprises de taille intermédiaire, qui sont essentielles à notre tissu économique et n'ont et n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation que les plus grandes. Nous saluons à cet égard, monsieur le secrétaire d'État, l'esprit de ce budget, qui, dans la lignée du précédent, vise à donner de l'air à nos entreprises et à faire de l'emploi la priorité. Nous aurons à coeur de contribuer à ce mouvement dans la discussion qui aura lieu dans les prochains jours. J'en viens à présent aux grands équilibres macroéconomiques et à la question de la dépense publique. Malheureusement, en 2019, le montant des économies reste très insuffisant. La réduction des déficits publics, par exemple, n'est pas satisfaisante.

Ce déficit alimente une dette publique abyssale, de l'ordre de 100 % du PIB, et qui ne cesse de se creuser ! Je cite le Haut Conseil des finances publiques La France n'aura pas encore amorcé, à l'horizon de 2019, la réduction de son ratio de dette publique au PIB, à la différence de la quasi-totalité des pays européens. Cette situation, dont vous avez largement hérité- j'en conviens -, est intenable. Elle met en péril notre souveraineté nationale. Nous n'allons pas non plus assez loin dans la maîtrise de la dépense publique, et nous restons le champion de l'Union européenne en la matière.

Ces facteurs risquent de perturber ce projet de budget au moment de son exécution et de vous mettre, à un moment ou à un autre, face à des choix difficiles. La réponse à cette difficulté est bien sûr plus d'efforts, plus d'efforts dès maintenant Plus d'efforts sur la dépense publique, tout d'abord : après avoir réalisé seulement la moitié de la réduction prévue pour 2018, vous limitez aujourd'hui vos ambitions à 0,4 point de PIB d'économies, soit à peine 10 milliards d'euros. C'est trop peu.

Le passé nous enseigne que ce type de promesse ne se tient pas davantage en fin de quinquennat qu'au début. Je dois néanmoins saluer la sincérité accrue de ce budget,

Un mot à présent des collectivités territoriales, alors que se déroule en ce moment même le Congrès des maires. Les maires que nous recevons, ici, au Sénat nous font part de leurs inquiétudes et de leurs attentes. Vous nous proposez une stabilité globale des dotations, ce qui est à mettre à votre crédit, après des années de diminutions draconiennes et indiscriminées. Mais cette stabilité cache, comme souvent, de grandes disparités selon les communes. Nous vous proposerons des amendements pour amortir la charge pour les communes les plus défavorisées. De plus, la hausse de la fiscalité sur le inquiétante pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, aura sans aucun doute un impact fort sur les budgets locaux et pour les maires bâtisseurs. Enfin, nous attendons des précisions sur le remplacement de la taxe d'habitation, qui tardent à venir. Je conclurai, mes chers collègues, en essayant de dissiper les caricatures que j'évoquais au début de mon propos. Nous ne croyons pas que vous opposiez les Français les uns aux autres au travers de ce budget, ou que vous choisissiez une catégorie plutôt qu'une autre.

Le Premier ministre a clairement dit qu'il avait entendu cette détresse. Nous sommes confiants dans le fait qu'il prendra des mesures fortes pour y répondre. Notre groupe est prêt à vous y aider. Sur la voie d'une transition énergétique pragmatique, sur la défense des PME et des ETI, sur la promotion de l'innovation à la française, sur le respect de l'autonomie des collectivités territoriales et de la ruralité, nous avons des propositions à vous faire pour améliorer ensemble ce budget. Le temps presse, et nous sommes collectivement responsables. C'est un enjeu de cohésion nationale, de cohésion territoriale et de compétitivité internationale. Faisons des débats autour de ce projet de loi de finances un exercice collectif, positif et pragmatique, au service de la France et des Français.

à l'égard de la parole et de l'action du Gouvernement paraissant particulièrement et durablement atteintes. Au moment de l'élection présidentielle, la confiance des ménages était mesurée à un elle s'effondre aujourd'hui à 94 ! Cette situation, couplée aux aléas pesant toujours plus sur l'environnement international, amène à s'interroger sur le scénario de croissance retenu, certes crédible, mais sans doute optimiste.

un maximum. En 2017, ce même jour, le ministre Darmanin promettait une stabilité de la dépense publique- une première, selon le cite : « Notre stratégie est donc de dépenser beaucoup moins et de cesser de faire de l'impôt le refuge de notre lâcheté, en réduisant au contraire les prélèvements obligatoires pour stimuler l'économie et le pouvoir d'achat ».

Les seules économies réalisées le sont par des mesures de sous-revalorisation de certaines prestations, notamment des retraites, pour un montant de 3,5 milliards d'euros tout de même. Une nouvelle fois, les retraités et les familles sont mis à contribution. Ce n'est pas glorieux On ne s'étonnera pas, dès lors, que, même en isolant les mesures temporaires et de périmètre, le déficit annoncé pour 2019 reste supérieur à ceux de 2017 et- incroyable -de 2016, et ce, monsieur le secrétaire d'État, malgré les effets de manche de vos premiers mois d'activité. Sans surprise, l'État continuera de porter la totalité du besoin en financement des administrations publiques, au détriment des administrations locales et de sécurité sociale, qui présentent, elles, des soldes positifs attendus à des niveaux respectifs En 2017, le ministre Darmanin annonçait que l'État prendrait sa part dans la baisse des dépenses, pour plus de 40 %. Là aussi, on en est loin ! En matière de pouvoir d'achat, malgré une communication du Gouvernement portant sur 6 milliards d'euros de baisse des prélèvements en faveur des ménages en 2019, l'Institut des politiques publiques et tous deux que, après une année blanche en 2018, les ménages bénéficieront d'un gain de pouvoir d'achat très limité en 2019. Le gain maximum sera de 1 % pour les plus riches, quand la légère augmentation pour les classes moyennes se fera au détriment des plus modestes. La réalité, monsieur le secrétaire d'État, c'est que votre orientation économique et budgétaire ne porte pas les fruits que vous en attendiez. Pour le dire de manière très triviale, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas Cela creuse les inégalités, sans offrir de compensations réelles à celles et ceux qui ont le plus besoin de l'État. Ces éléments de contexte étant rappelés, je souhaite évoquer le volet recettes du projet de loi de finances pour 2019. 2019. Comme vous le savez, les parlementaires socialistes des deux chambres ont travaillé sur une proposition alternative de budget pour la France et pour les Français. Nous le disons ici avec force, nous pouvions dégager davantage de recettes

de recettes. Nous sommes contre la suppression de l', que vous envisagez. Nous sommes contre l'élargissement de la « niche Copé », que vous nous soumettez.

Vous auriez pu ainsi éviter la vente d'actions, notamment celles d'Aéroports de Paris, proposée dans le même projet de loi. Quand ces mesures se doublent d'un accroissement de la CSG personnalisées au logement, les APL, de coupes opérées au détriment de nos territoires périphériques- je pense en particulier aux outre-mer, qui subissent un traitement très dur dans ce projet de loi de finances -ou encore d'une désindexation

l'examen du PLFSS, d'appliquer la revalorisation initialement prévue des pensions du régime général, de corriger la hausse de la CSG en ne l'appliquant qu'aux pensions les plus élevées ou encore de mettre en place un minimum vieillesse de 85 % du SMIC pour les retraités agricoles. C'est pourquoi, nous souhaitons accélérer la transition énergétique de l'économie française, vos actions n'étant pas suffisantes à nos yeux, comme en attestent, à la fois, le projet de loi de finances rectificative pour 2018, que nous venons d'examiner, et le projet de loi de finances pour 2019. Notre collègue Rémi Féraud interviendra plus précisément sur ce point majeur, sur lequel l'attention est particulièrement focalisée aujourd'hui. aujourd'hui. Parce que vous ne faites pas assez en faveur de la cohésion sociale, il convient de mettre de toute urgence en place des actions en ce sens. Notre pays doit absolument s'engager dans une nouvelle manière de penser la prise en charge de nos aînés.

au logement au regard de l'inflation, contrairement à ce qui est proposé dans le présent texte. Certes, cette orientation n'est pas compatible avec la « start-up nation » prônée par le Président de la République, mais notre pays n'est pas une entreprise. C'est une communauté de destin, en droit d'attendre davantage de considération de leurs responsables politiques. Durant l'examen de ce texte, nous formulerons plusieurs propositions par voie d'amendements.

par une paupérisation accrue des classes populaires et que les ressources supplémentaires servent réellement à financer la transition écologique et énergétique. Concrètement, cela se traduit par un élargissement de l'assiette de la taxe d'enlèvement des

En seconde partie, nous évoquerons également la question du chèque énergie, à la lumière des dernières annonces du Gouvernement. En matière environnementale, nous allons proposer la suppression de la fiscalité réduite pour les produits à base d'huile de palme. Il s'agit vraiment d'une anomalie, qu'il convient de corriger.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, certes, le contexte que nous connaissons cette année et dans lequel nous allons devoir examiner ce projet de loi de finances, est radicalement différent de celui que nous avons connu l'an passé, au moment de l'examen du budget de l'année qui s'achève.

On ne peut pas se plaindre, sans cesse, de l'instabilité fiscale, des changements de pied permanents, et critiquer le fait qu'un projet de budget soit en cohérence avec le précédent

la trajectoire décidée par le Gouvernement plonge actuellement le pays dans une grave crise. Je ne crois pas que cette crise soit due exclusivement, ni même principalement, à la fiscalité écologique. Celle-ci, certes mal calée, est victime de l'ensemble de la politique gouvernementale, de son injustice fiscale, manifeste depuis dix-huit mois, comme des promesses non tenues en matière de pouvoir d'achat.

Mais quelle erreur de l'avoir à ce point dissociée de son impact social ! Très bien ! C'est l'élu parisien qui vous le demande, monsieur le secrétaire d'État : comment accepter l'idée que cette fiscalité frappe essentiellement ceux qui vivent en milieu rural, avec de longues distances à parcourir et, surtout, et, surtout, sans moyens de transport alternatifs plus écologiques sur lesquels se reporter ? En l'absence de véritable mesure compensatoire à l'égard des ménages modestes les plus dépendants aux énergies fossiles, les mesures prises pénalisent de manière particulièrement dure et injuste leur pouvoir d'achat.

C'est une attitude dangereuse, car elle renforce les frustrations- nous le voyons bien ces jours-ci -et, par conséquent, elle risque de mettre en danger la notion même de fiscalité écologique. Très bien ! C'est d'autant plus aberrant que de nombreuses pistes peuvent être ouvertes pour répondre au mécontentement qui s'exprime.

Contrairement à un gel complet ou à un moratoire durable, cela ne remettrait pas en cause la volonté d'aller vers un bilan carbone neutre de notre pays en 2050, mais permettrait de prendre en compte la hausse actuelle du prix du pétrole, de se donner le temps, dans les années à venir, de mieux répartir les efforts et de repenser les mesures d'accompagnement en faveur des ménages particulièrement pénalisés.

permettrait de rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangés par l'État du fait de la hausse des cours du pétrole, comme l'avait fait le gouvernement Jospin en 2001. Nous proposerons un amendement dans ce sens on nous répondra que son effet serait minime. Dès lors, pourquoi le refuser par principe ? Par ailleurs, et c'est le point essentiel, nous considérons que les recettes des taxes sur l'énergie devraient être intégralement redirigées vers des actions en faveur de la transition énergétique. C'est certainement là que le bât blesse le plus. Rien de tel n'est fait, comme le montre encore le reversement de 600 millions d'euros de recettes de TICPE vers le budget général de l'État, marque d'une absence de volontarisme total en matière de transition énergétique. C'est un mauvais signal envoyé, car tout ce qui contribue à faire de la taxe carbone une taxe de rendement budgétaire lui fait perdre de sa légitimité. De nombreuses pistes d'amélioration des politiques publiques existent, comme l'aide à la rénovation thermique, à l'isolation des logements, l'augmentation de la prime à la conversion automobile- une aide à laquelle le Gouvernement se convertit lui-même lentement -, sans parler de la nécessité, dans cette période transitoire, d'apporter un soutien financier aux plus modestes pour payer leurs factures de chauffage ou de carburant. Enfin, je profite de cette intervention pour renouveler notre proposition, très largement partagée, d'une conférence nationale sur le financement de la fiscalité écologique, afin de sortir par le haut, et avec tous les partenaires concernés, de la crise actuelle et de l'impasse dans laquelle s'est mis le Gouvernement. Car la fiscalité écologique n'est pas isolée. Au contraire, elle devrait être une composante de la lutte contre les inégalités. Il n'est plus possible de concevoir séparément politique environnementale et politique sociale. Pour notre part, au groupe socialiste et républicain, nous pensons que cette transition énergétique est une bataille collective, qu'elle ne peut se gagner que dans le cadre d'un contrat social juste et donc accepté par les Français. Nous avons la conviction que c'est possible si la volonté politique est là.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2019 s'inscrit encore cette année dans une trajectoire de maintien du déficit public sous la barre des 3 %, conformément à notre engagement européen. Constaté à 2,7 % en 2017, attendu à 2,6 % en 2018 et espéré à 2,8 % pour l'année prochaine, avec un tel taux, tant bien que mal, la France reste dans les clous. La procédure pour déficit excessif a été levée, mais elle demeure comme une épée de Damoclès si le scénario de croissance le plus défavorable venait à faire basculer notre déficit à 3,2 %. C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure compte tenu du contexte international, qui génère, vous serez d'accord avec moi, quelques incertitudes. Notre collègue rapporteur de la commission l'a souligné : l'hypothèse de croissance à 1,7 % est bien fragile, sous l'effet notamment de la remontée des prix du pétrole, des menaces de guerre commerciale régulièrement brandies par le dirigeant américain, ou encore du Brexit, dont on ne mesure pas encore l'impact sur l'économie européenne. En attendant, la crédibilité budgétaire de notre pays doit être consolidée. Le Gouvernement, c'est vrai, s'y emploie, sous la pression de la Commission européenne, mais aussi du Haut Conseil des finances publiques, qui exerce un rôle de vigie bienvenu, pour ne pas dire bienfaiteur. Pour autant, les résultats, nonobstant cette volonté de rétablissement d'une trajectoire plus saine de nos finances publiques, ne sont pas encore suffisants. Le déficit augmente l'an prochain, mais il est vrai que le reclassement de la dette de la SNCF au sein des administrations publiques pèse lourd, très lourd. L'effort de maîtrise des dépenses publiques est quelque peu écorné, puisque celles-ci devraient croître de 0,6 % en volume. Par conséquent, le déficit structurel peine à se résorber. L'embellie budgétaire dépend trop de la dynamique conjoncturelle. Le déficit structurel, en réalité, est notre vraie faiblesse au regard des règlements européens et il déclasse la France par rapport à nos partenaires, au premier rang desquels figure l'Allemagne, bien entendu. Il faut toutefois reconnaître que l'exercice n'est pas facile, d'autant que l'on ne peut pas ignorer le caractère encore prégnant d'un héritage qui, n'ayons pas peur de le dire, est à mettre au compte de tous les gouvernements qui se sont succédé. En effet, comment, mes chers collègues, faire table rase de quarante-cinq de budgets déficitaires ? Dans ces conditions, la dette de la France sera de 98,7 % du PIB pour l'année prochaine, un niveau très élevé. Au sein de la difficile équation entre baisse des dépenses et coup de pouce à l'activité, le Gouvernement a fixé des priorités, dont certaines, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas bien comprises. Je pense bien sûr à la question des impôts et taxes affectant nos concitoyens, qui a conduit plusieurs milliers d'entre eux à exprimer leur ras-le-bol fiscal dans la rue. C'est préoccupant, car le consentement à l'impôt-

que ce soit la suppression des cotisations chômage ou le dégrèvement de la taxe d'habitation. Mais il existe un décalage entre la mise en oeuvre des dispositifs et les effets qu'ils produiront à plus ou moins long terme. L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, vient de rappeler que le revenu disponible des ménages avait baissé en moyenne de 440 euros entre 2008 et 2016. 2016. Pour le moment, c'est cette réalité que vivent nos concitoyens et il faudra peut-être réorienter certains dispositifs fiscaux touchant au pouvoir d'achat, avec plus de mesure, comme le propose d'ailleurs la commission des finances. S'agissant du verdissement de la fiscalité, qui alimente une partie des hausses des carburants, si elle doit s'exercer au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, cela ne peut pas être fait avec brutalité, mais aussi sans équité.

Pour ma part, j'y souscris, car cela va dans le sens d'un allégement du coût du travail évidemment nécessaire dans ce monde de plus en plus ouvert que nous connaissons. je souhaitais souligner l'importance de soutenir plus directement l'industrie, dont le décrochage est alarmant : elle ne représente actuellement plus que 12,4 % du PIB, contre 16,5 % dans les années 2000. l'industrie est un puissant vecteur de soutien des bassins d'emploi et de dynamisme des territoires. L'impact de la transformation du CICE sera-t-il à la hauteur pour des secteurs exposés à la concurrence internationale, sachant que le dispositif est centré sur les bas salaires ? je voudrais rebondir sur vos propos concernant les chantiers à poursuivre au sein de l'Union européenne. On doit en effet tout mettre en oeuvre pour éviter une concurrence intra-européenne qu'alimente un certain social. Amazon -ou l'union des marchés de capitaux sont quelques-uns des outils qui donneront plus de sens à la solidarité européenne : on ne peut pas, d'un côté, imposer des règles budgétaires vertueuses, et, de l'autre, laisser perdurer la non-coordination des politiques fiscales européennes. Voilà quelques remarques que je souhaitais faire au nom du RDSE sur ce projet de loi de finances, qui, je l'espère, sera enrichi au fil de nos débats.

collègues, lors de la présentation de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a fixé des objectifs à court et moyen terme. Je voudrais à cet instant revenir sur plusieurs de ses engagements et les examiner au regard du projet de loi de finances pour 2019. Sur l'assainissement de nos finances publiques, monsieur le secrétaire d'État, vous aviez fixé un cap pour la durée du quinquennat : moins 5 points de dette publique, moins 3 points de dépense publique, moins 1 point de prélèvements obligatoires.

le ciel conjoncturel, notamment avec le ralentissement de la croissance, pensez-vous, monsieur le secrétaire d'État, pouvoir tenir le cap, atteindre les objectifs fixés et gagner ce pari difficile, mais nécessaire, du redressement de nos comptes publics ? de votre engagement à gagner le pari de l'emploi, après tant d'efforts sincères faits par les gouvernements successifs sans résultat probant, après tant de mesures qui n'ont pas abouti à mettre en échec le chômage de masse, vous avez souhaité ouvrir une nouvelle voie en faisant le pari de réussir à endiguer le chômage par une meilleure compétitivité de nos entreprises, l'allégement de leur fiscalité, l'allégement de la fiscalité du capital, la relance de l'investissement. Cette année, vous prolongez cette ligne en concrétisant la bascule du CICE en allégements de charges, en poursuivant la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, en adaptant la fiscalité des petites et moyennes entreprises aux défis de la nouvelle économie et de la robotique, également par la modernisation de la fiscalité agricole ou encore par la mise en oeuvre du volet fiscal de la loi PACTE, qui devrait par exemple faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises. Comme je l'avais indiqué l'an passé, nous voulons bien vous accompagner sur cette nouvelle voie en faveur de l'emploi, là où tant d'autres politiques ont échoué, à condition qu'il y soit prévu des mesures concrètes pour réduire les inégalités, afin de ne pas fragiliser les plus démunis

tant ils accompagnaient utilement les plus démunis et contribuaient à l'offre de services, notamment dans le secteur associatif. Nous le savons bien, les effets de vos choix en matière d'emploi ne peuvent pas donner leur pleine mesure immédiatement, mais les résultats devront néanmoins être au rendez-vous d'une baisse significative et durable du chômage. Quelles sont vos prévisions en la matière ? Quand verra-t-on, selon vous, les effets de vos choix politiques et, donc, une baisse du chômage en France ? Autre sujet d'actualité, s'il en est : la transition énergétique. Celui-ci est trop important pour qu'on sombre dans le déni ou la démagogie. Nous sommes en train de détruire notre planète. Voilà la réalité ! Les conséquences, nous les connaissons et elles sont alarmantes. Peut-on continuer ainsi ? Peut-on expliquer à nos enfants que c'est l'héritage qu'on veut leur laisser ? Aucun d'entre nous ne le pense, et donc nous devons l'assumer en responsabilité : les énergies fossiles ne peuvent pas être l'avenir. Nous devons donc réduire notre consommation d'énergies fossiles et accélérer le passage à d'autres sources d'énergie, accélérer aussi l'utilisation dans nos pratiques industrielles, agricoles et individuelles de produits respectueux de l'environnement et de la santé publique. Nous devons changer nos comportements. Mais les mesures incitatives, les taxes incitatives, pour être acceptées, doivent être comprises ; pour être comprises, elles doivent être justes. ! Pour cela, il faut, premièrement, qu'il existe une solution de remplacement, et, deuxièmement, quand cette autre solution existe, qu'elle soit financièrement accessible pour tous. C'est bien le problème aujourd'hui : monsieur qui êtes élu d'un département en partie rural, comme le mien, dites-moi comment faire accepter une hausse de taxes incitative aux habitants des milieux ruraux lorsqu'ils n'ont pas d'offre alternative pour se déplacer ? Comment faire accepter une hausse du prix du fioul aux familles à revenus modestes, qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer le changement de la chaudière au-delà du crédit d'impôt, certes significatif, mais qui ne couvre que 30 % de l'opération ? Monsieur le secrétaire d'État, je le dis en responsabilité : nous devons garder l'objectif d'une accélération de la transition énergétique, il faut garder le cap, c'est notre responsabilité de l'expliquer, et rien ne serait plus irresponsable que de prétendre le contraire, mais, pour réussir, il faut accélérer la mise sur le marché de solutions alternatives, il faut renforcer les mesures d'accompagnement, il faut revoir la trajectoire de la hausse. Très bien ! Tout à fait d'accord ! Enfin, je voudrais évoquer rapidement deux autres sujets. de la fiscalité agricole, je tiens à saluer le travail qui a été mené en étroite collaboration avec la profession et un groupe de parlementaires auquel vous avez bien voulu m'associer. L'agriculture joue un rôle primordial dans l'économie de notre pays, et elle joue aussi, ne l'oublions jamais, un rôle majeur dans l'aménagement du territoire en faisant vivre la ruralité. Le dispositif d'épargne de précaution plus ouvert et plus souple, le relèvement du plafond pour faciliter la transmission des baux ruraux, la possibilité de revenir sur son choix de régime fiscal ou encore le maintien du régime du micro-BA, bien adapté aux exploitations de petite taille et très pratiqué en zone de montagne, sont autant d'avancées que je tiens à saluer. S'agissant des collectivités locales,

mesures étaient nécessaires, d'autres non -, il y avait besoin de stabilité et de lisibilité. Vous avez apporté dès 2018 cette stabilité, tant dans le montant des dotations que dans l'organisation territoriale. C'était nécessaire. Pour 2019, le maintien de la DGF à son niveau de 2018, la hausse de la péréquation ou encore la réforme de la dotation d'intercommunalité, qui revient sur le dispositif injuste des catégories d'EPCI, vont dans le bon sens, de même que la péréquation à destination des départements ayant le plus de difficultés à faire face aux dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité. Toutefois, la réduction des crédits affectés aux contrats de ruralité,

Une remise à plat est aujourd'hui nécessaire et j'ai compris que le Gouvernement était prêt à engager ce chantier. Enfin, nous suivrons avec la plus grande attention le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale, qui devrait être examiné au printemps prochain. La commission des finances a d'ores et déjà fait des propositions concrètes à ce sujet. La parole

je vais, comme l'an dernier, utiliser mon temps de parole pour évoquer la politique du logement du Gouvernement et ses conséquences, qui se dessinent maintenant très nettement, mais aussi pour parler de nos collectivités territoriales, acteur majeur du secteur. d'État, les prévisions sur lesquelles vous vous êtes fondés pour construire ce budget paraissaient prudentes. Vous aviez d'ailleurs ramené votre prévision de croissance à 1,7 %. En matière de logement, l'année s'annonçait en retrait par rapport à 2017, mais vous étiez encore rassurants.

Mais voilà, depuis lors, le ciel s'est sérieusement assombri. Conséquences de la guerre commerciale de M. Trump, de la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis et du prix du pétrole, des incertitudes liées au Brexit la croissance ralentit- le consensus est maintenant à 1,6 % -, le chômage ne baisse pas, ou si peu, le moral des Français est en berne et l'investissement industriel également. Il y a cependant un secteur d'activité qui aurait pu se trouver relativement à l'abri de ces turbulences, en tous les cas tant que les taux d'intérêt restent sages : il s'agit du logement. Malheureusement, c'est la cible principale que vous avez choisie l'an dernier

Ce n'est pas faute d'avoir, l'an dernier et en juillet encore, lors de la discussion de la loi ÉLAN, attiré votre attention sur le risque que vous faisiez courir à un secteur qui sortait à peine du marasme des années 2014 et 2015. Mais au fait, comment ce marasme a-t-il été déclenché à

Eh bien voilà, nous y sommes, et malheureusement bien plus vite que prévu ! L'année 2018 s'annonçait en effet en net repli, alors même qu'il y a, dans le secteur, un retard inhérent à l'inertie des projets.

et les professionnels du bâtiment parlent maintenant de 120 000 emplois en jeu dès l'année prochaine, et potentiellement de 200 000 emplois à l'horizon 2020. Allez-vous au moins, au nom du Gouvernement, reconnaître que ces chiffres sont conformes à la réalité ? Je vous pose la question puisque, jusqu'à présent, le Gouvernement a été dans le déni absolu. Ce n'est plus possible. Si vous reconnaissez que ces chiffres sont exacts, il faut en tirer les conséquences dès maintenant ! Si j'en juge le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, la réponse est malheureusement non. C'est même exactement le contraire, avec deux mesures figurant dans le texte initial du Gouvernement

Ce n'est que par voie d'amendement que le Gouvernement a desserré- mais si peu -le dispositif Pinel dans le cadre des opérations Coeur de ville et accepté le retour de l'APL accession, mais seulement dans certains territoires d'outre-mer. Ce n'est pas avec ces mesures, monsieur le secrétaire d'État, que vous inverserez la tendance. Il faudrait, selon nous, revoir d'urgence le zonage, ce qui aurait déjà dû être fait, car il ne permet pas de cibler correctement les aides fiscales. Il faut rétablir l'APL accession sur tout le territoire : cela ne coûterait que 50 millions d'euros de plus l'an prochain et ce serait parfaitement cohérent avec votre objectif de vente d'HLM. Il faut recalibrer le PTZ pour soutenir l'accession à la propriété partout. Monsieur le secrétaire d'État, si vous ne voulez pas prendre le risque d'une crise majeure dans le secteur, il faut bouger maintenant.

allons vers une véritable réforme de la fiscalité du secteur, mais, d'ici là, il faut des mesures pour soutenir celui-ci et éviter son effondrement. S'agissant des bailleurs sociaux,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, à mon sens, nous ne pourrions terminer cette discussion générale sans évoquer de nouveau la situation explosive sur l'île de la Réunion, été question au cours des questions d'actualité. J'exhorte vraiment le Gouvernement à y accorder une importance et un soin particuliers,

J'espère qu'on saura trouver les voies et les moyens pour engager des discussions et arriver à un accord un peu plus global. En 2017, nous avons tous été attentifs aux mots du Président de la République, d'abord dans ses écrits de candidat, puis lors de la campagne, ensuite dans son fameux discours de Versailles. Ses mots étaient « girondisme », respect de l'autonomie des territoires », « respect des élus », « progrès social », « justice fiscale ». Deux ans après, la déception est grande. Partout en France, comme mes collègues et moi, monsieur le secrétaire d'État, vous entendez monter et gronder la colère. Celles et ceux qui ont fait confiance ne cessent, disons-le, de dévisser et ce budget n'est pas de nature à opérer une reconquête des coeurs et des esprits. Comme moi, vous entendez sûrement le peuple et les élus dénoncer la rigidité et la brutalité du pouvoir ; vous entendez ceux qui dénoncent- eh oui ! -le mépris, l'arrogance, voire la vanité. L'impression tenace, c'est celle d'une absence d'humanité et d'une faute de coeur. Bien sûr, tout cela est peut-être surjoué, mais l'intelligence politique commande de tenir compte du vécu et du ressenti des populations. Mes chers collègues, pour illustrer l'écart entre les promesses et les réalités, j'aimerais pouvoir vous exposer, vous expliquer les « mauvaisetés » infligées aux outre-mer. Pour les outre-mer, le candidat Macron s'était engagé sur plus de 4,5 milliards d'euros : 1 milliard d'euros dans une lettre publiée opportunément par l'hebdomadaire en Nouvelle-Calédonie, que tous les électeurs ont reçue

faite de verticalité raide, d'expertise aveugle et technocratique, d'indifférence brutale, si ce n'est de mépris affiché pour les élus, comme s'ils ne pouvaient être de bons experts de la situation de leur population et de leur territoire.

ainsi que les socioprofessionnels de nos territoires, lorsqu'il s'est agi de préparer la réforme des aides économiques outre-mer ? Était-il utile d'organiser les assises des outre-mer, alors même que, dès janvier, nous connaissions les arbitrages de l'État ? C'était une belle entreprise de communication ! Tout cela nous a fait perdre deux ans pour, finalement, aboutir à une réforme de pur rendement, pensée par vos services et prétendument légitimée par les conclusions de ces assises. Est-il fiscalement juste de proposer une augmentation frénétique,

efficace de supprimer les outils permettant de construire des logements sociaux ou de mettre fin aux dispositifs favorisant le développement des zones géographiques les plus défavorisées ? Puisque j'ai épuisé mon temps en disant au Gouvernement que le Sénat a une culture du compromis raisonnable et intelligent. Nous tenterons, après un travail transpartisan, de proposer des solutions raisonnables. J'espère,

de loi de finances pour 2019 comporte peu de mesures très importantes relatives aux collectivités territoriales. Le Gouvernement a annoncé pour le printemps 2019 une loi de finances rectificative qui abordera notamment l'épineuse question de la réforme de la taxe d'habitation, laquelle représente, je le rappelle, un tiers des recettes fiscales du bloc communal. En effet, la suppression de cette taxe pour 100 % des ménages, imposée par le Conseil constitutionnel, interviendra en 2021, si j'en crois les propos tenus par le ministre Gérald Darmanin lors de la discussion du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. La suppression totale de la taxe d'habitation fera peser sur les finances publiques une surcharge de près de 14 milliards d'euros en 2020 par rapport à la trajectoire inscrite dans la loi de programmation des finances publiques, surcharge qui sera financée par le déficit. Ainsi, l'allégement d'impôt pour le contribuable local sera financé par le contribuable national ... Au cours des débats à l'Assemblée nationale,

ainsi qu'à votre cabinet et aux équipes de Bercy, bien du courage pour traiter tous les problèmes soulevés dans un laps de temps aussi court ! Le premier semestre de 2019, c'est demain. Si cette loi doit être le Grand Soir de la fiscalité des collectivités locales, je m'étonne que le projet de loi de finances pour 2019 comprenne un certain nombre de dispositions faisant évoluer de manière autonome des dispositifs existants : réforme de la dotation d'intercommunalité, à l'article 79, modification des modalités de répartition de la dotation politique politique de la ville, à l'article 81, transformation de la dotation globale d'équipement des départements en une dotation de soutien à l'investissement départemental. L'étude d'impact annexée au projet de loi ne donne aucune simulation de ces évolutions. Tout au plus sait-on que « la modification des règles de plafonnement de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des départements est neutre pour la catégorie des départements et n'a d'effet qu'au niveau individuel » ou encore que « la réforme de la dotation d'intercommunalité d'intercommunalité est neutre pour la catégorie des EPCI à fiscalité propre et n'a d'effet qu'au niveau individuel ». Il n'était pas besoin d'étude d'impact pour écrire cela ... Nous aurons très certainement de riches débats sur la réforme de la fiscalité locale au printemps prochain. Il est cependant certain que nous ne pourrons continuer à légiférer en empilant des dispositifs sans aucune simulation à maille fine. C'est toujours le problème. Par ailleurs, en tant que sénateur des Hauts-de-Seine, je ne peux que rappeler l'impatience des élus franciliens quant à une prise de décision sur l'organisation institutionnelle de la région d'Île-de-France. Le millefeuille à cinq couches est indigeste En tant que sénateur du groupe Les Républicains, je veillerai à ce que le nouveau système fiscal proposé préserve la libre administration et l'autonomie financière des collectivités locales. Pour en revenir au projet de loi dont nous allons débattre ces prochains jours, 11 des 85 articles du texte initial concernent directement les finances locales. Conformément à l'engagement pris en 2017 de ne pas diminuer les dotations aux collectivités en contrepartie de la mise en oeuvre du dispositif de contractualisation, l'article 23 maintient le niveau de la dotation globale de fonctionnement pour 2019 à son niveau de 2018. Ce maintien en euros courants masque cependant une baisse en euros constants dès lors que l'inflation repart à la hausse.

Il aurait donc été de bon ton que l'État respecte le sien. Ce qui est vrai en général- le maintien des dotations -est faux en particulier : en 2018, près de la moitié des communes ont vu leur DGF diminuer et les deux tiers ont été touchées par une baisse de leur dotation forfaitaire. En effet, afin de respecter les plafonds fixés par l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 en ce qui concerne la trajectoire des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, toute hausse doit être gagée par le biais des variables d'ajustement. Ainsi, en 2019, les variables d'ajustement sont minorées à hauteur de 144 millions d'euros. Selon le Gouvernement, « les variables d'ajustement relatives à chaque catégorie de collectivités doivent neutraliser les hausses de crédits gagées qui lui bénéficient » ; dit autrement, cela revient à donner d'une main pour reprendre de l'autre, ou encore à à financer de la péréquation verticale par de la péréquation horizontale. Cette année, cette logique n'est pas parfaitement respectée, puisque le bloc communal viendra financer à hauteur de 34 millions d'euros l'augmentation des ressources des départements. La loi de finances pour 2018 avait élargi l'assiette des variables d'ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes et des En avril 2018, une instruction fiscale de Bercy venait geler l'application de cette disposition pour les EPCI, au regard de sa très forte concentration. Les mêmes effets se sont fait sentir lors de la ventilation de la minoration sur les communes, conduisant même quatre maires des Hauts-de-Seine à attaquer en justice l'arrêté préfectoral de notification.

Je rappellerai simplement que le parc automobile des collectivités territoriales est composé à hauteur de 75 % par des véhicules diesel. Je citerai également l'augmentation des tarifs de la composante « déchets » de la TGAP entre 2021 et 2025. Bien évidemment, les apporteurs de déchets doivent être incités à privilégier les opérations de recyclage. Cependant, comme 30 % des déchets des ménages ne sont aujourd'hui

sur le gazole non routier, le GNR, va pénaliser à hauteur de 500 millions d'euros le secteur des travaux publics ; il ne vous aura pas échappé que ce surcoût sera très certainement refacturé aux clients. Or les donneurs d'ordres en matière de travaux publics sont à hauteur de 65 % les collectivités

proximité AMF-CEVIPOF : « la recentralisation ressentie de l'action communale ne se traduit pas par le transfert de compétences communales à l'État central, mais résulte plutôt des contraintes budgétaires installées dans la durée ».

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, un budget, c'est d'abord des visages, des personnes, des enfants dont nous cherchons à améliorer la vie. Ces visages, ce sont d'abord pour moi ceux des Français de l'étranger, que je représente ici avec d'autres. évoquer les conséquences fiscales de ce projet de budget pour nos compatriotes expatriés. Le Gouvernement décrit comme une conquête sociale la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des Français. Cela ne concerne pas, évidemment, les Français de l'étranger qui ont une résidence en France. Il serait intéressant de savoir quand les Français de l'étranger pourront enfin obtenir que leur résidence unique en France soit considérée comme leur résidence principale. Bercy a lâché du lest sur quelques impôts dans ce projet de budget, en matière de plus-values ou de pensions alimentaires notamment, mais on reprend d'une main ce que l'on a accordé de l'autre. Le taux minimum d'imposition sur les revenus de source française augmente de 20 % à 30 %. J'ai déposé un amendement de suppression de cette augmentation. Nos compatriotes m'écrivent pour s'inquiéter de la mise en oeuvre du prélèvement à la source. Ils ont le sentiment que le nouveau système leur sera défavorable et qu'ils paieront davantage. Aux questions écrites que j'ai posées à ce sujet, vous avez répondu, monsieur le secrétaire d'État, qu'il n'y aurait pas un double prélèvement. Mais que se passera-t-il quand existe une convention fiscale ? Le prélèvement à la source sera-t-il, dans ce cas, opéré sur les revenus de source française ? En matière de CSG-CRDS, nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne ont été exonérés, mais les autres Français résidant dans des pays tiers sont restés sur leur faim. Pourquoi celui qui vit en Belgique, en Italie ou en Espagne serait-il exonéré de la CSG-CRDS, et pas celui qui vit en Chine, aux États-Unis, en Afrique ou en Australie ? Où est l'« égalité » qui figure dans notre belle devise ? outre, on n'a dispensé personne de la nouvelle contribution de solidarité de 7,5 %. En ce qui concerne notre réseau scolaire à l'étranger, le Président de la République a prévu le doublement du nombre d'élèves d'ici à 2030. Il s'agit de faire toujours plus avec des moyens qui soit diminuent, soit stagnent. du nombre d'élèves suppose pratiquement un doublement du nombre d'enseignants. Or le gouvernemental, c'est la stabilisation des moyens et la réduction des effectifs, alors que les besoins augmentent. Par quel exercice de prestidigitation allez-vous réaliser ce programme ? à l'étranger, l'AEFE, est stable. Elle est fixée à 384 millions d'euros. Pour compenser les conséquences de la suppression de 33 millions d'euros de crédits l'an dernier, l'AEFE a porté unilatéralement son prélèvement sur les établissements conventionnés de 6 % à 9 %

Au lieu de modifier le barème des bourses alors que les besoins des familles augmentent, on bloque le système en réduisant la dotation de l'État, et on fragilise l'AEFE. En 2017, les parents ont participé à hauteur de 65 % au financement des établissements en gestion directe et des établissements conventionnés. Le Président de la République a indiqué qu'une des solutions qu'il préconisait était la recherche de partenariats locaux ou de mécénats. Toutefois, cette recherche se révèle complexe et aléatoire et ne permet pas d'avoir une véritable visibilité pour un fonctionnement sain et pérenne des établissements scolaires.

La législation ne permet plus de renouveler un CDD au-delà de six années, et le ministère remercie des agents qualifiés et expérimentés pour les remplacer par de nouvelles recrues qui n'auront évidemment pas la même expérience et les mêmes qualifications. On marche sur la tête

Bref, encore une fois, les Français de l'étranger sont pénalisés : hausse du taux minimum d'imposition sur le revenu de 20 % à 30 %, instauration d'une taxe de solidarité, réduction des budgets des postes diplomatiques, réduction des subventions à l'AEFE, diminution des bourses Mais quel est votre problème avec les Français de l'étranger ? Ils sont avant tout français, et nous sommes fiers de leur courage. Ils ont droit à notre considération et à votre attention. Ne pensez pas à eux uniquement au moment des élections, car ils ont de la mémoire et sauront se souvenir de la manière dont ils ont été traités

et accompagner la création d'emplois, grâce au renforcement des mesures d'allégement qui avaient déjà été programmées et à la mise en place d'un nouvel allégement en remplacement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

à compter de l'automne prochain et la suppression du forfait social à la fois sur l'intéressement et la participation, selon la taille des entreprises. Ces mesures sont financées

ce projet de loi de finances, ce sont plus de 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat que nous rendons aux ménages, avec, il est vrai, 3 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire, dont une partie est liée à la fiscalité écologique- j'y reviendrai dans un instant -, mais surtout 9 milliards d'euros d'allégements,

Les dépenses de l'État pour la norme pilotable baisseront de 0,5 % en volume en 2019, soit une augmentation en valeur de 0,8 %. Il faut rapporter ces chiffres à la hausse de 2,3 % des dépenses locales, investissement et fonctionnement compris, ou à celle de 2,5 % des dépenses d'assurance maladie.

D'ailleurs, ce n'est pas à une assemblée parlementaire que j'apprendrai que le principe d'universalité budgétaire interdit la généralisation des affectations de ressources. Sinon, nous aurions non plus une loi de finances, mais un simple empilement de comptes d'affectation spéciale. Le principe de la fiscalité comportementale que nous mettons en oeuvre est de décourager la consommation de produits nocifs pour notre santé ou notre environnement, et non pas de financer des dépenses nouvelles. Telle est la philosophie qui est la nôtre en matière de fiscalité écologique. Le Premier ministre a annoncé récemment de nouvelles mesures d'accompagnement,

De même, le chèque énergie sera porté de 150 euros en moyenne à 200 euros par an, ce qui représente un engagement budgétaire de 740 millions d'euros, contre 560 millions d'euros

suite des assises des outre-mer, la ministre des outre-mer a en effet pris, monsieur Lurel, des décisions courageuses au bénéfice direct des territoires ultramarins : la suppression de la TVA-NPR,

Ils s'élevaient à 47,8 milliards d'euros en 2017, à 48,1 milliards d'euros en 2018 et ils sont fixés à 48,2 milliards d'euros dans le projet

le premier relève de l'écrêtement de la dotation forfaitaire pour financer des emplois internes, notamment en matière d'augmentation de la péréquation verticale ; le second tient au fait que la DGF est aussi allouée aux communes, notamment pour ses parts péréquées- la DSU, la DSR et, souvent, la DSR « cible » -, selon leur potentiel financier agrégé. Le potentiel Le potentiel financier agrégé tient compte d'indicateurs socio-économiques propres à la commune, mais aussi à l'intercommunalité d'appartenance. La modification importante de la carte intercommunale intervenue au 1 janvier 2017 a, d'une manière

À critères constants, l'année 2019 s'annonce sous de meilleurs auspices, pour une raison très simple : la carte intercommunale a extrêmement peu bougé au 1 janvier 2018. Ainsi, le potentiel financier agrégé de référence

En 2018, elles s'établissaient à 323 millions d'euros, dont ont été retranchés, par décision de gestion, environ 120 millions d'euros au titre de la DCRTP des intercommunalités, que Gérald Darmanin et moi-même avons décidé de ne pas minorer après l'adoption du projet de loi de finances pour 2018. Nous sommes aujourd'hui à 144 millions d'euros.

Le Président de la République a dit hier, devant les maires réunis à l'Élysée, qu'il était favorable à un débat sur les modalités de répartition, tout en soulignant combien il était difficile d'aboutir à une solution qui satisferait tout le monde, sachant que l'enveloppe est normée et que les marges de manoeuvre budgétaires sont relativement contraintes.

une ressource qui soit pérenne, juste et durable. Nous aurons à travailler, dans les prochaines semaines, sur de nouvelles modalités de répartition du fruit des impôts locaux. Nous devrons préciser ce qui doit être compensé parce que supprimé et ce qui ne sera pas compensé parce que non supprimé. Nous avons d'ores et déjà indiqué la volonté du Gouvernement

Cela nous permettra d'ouvrir un débat sur la manière dont les collectivités territoriales et l'État pourront continuer à percevoir un certain nombre de taxes ou d'impôts : je pense à la contribution pour le financement de l'audiovisuel public, à la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou encore à la taxe spécifique et facultative mise

L'article liminaire du projet de loi de finances pour 2019 appelle évidemment quelques observations. Il convient, à tout le moins, de relever les mouvements affectant notre système de prélèvements. Sans même parler du sentiment profond des Françaises et des Français au regard de l'impôt, force est de constater que l'année 2019 est marquée par une double rupture.

Le journal nous apprend aujourd'hui que seulement 54 % de nos concitoyens jugent le paiement de l'impôt comme un acte citoyen. À force de fragiliser l'impôt dans le discours politique,

à la compensation des allégements de cotisations sociales, aux droits sur les tabacs, alcools, bières, cidres, etc., ressources d'ores et déjà transférées pour boucher les trous de la sécurité La fiscalisation de la sécurité sociale préfigure sans doute l'activation d'un nouveau système, visant à affecter les éventuels excédents de comptes sociaux au comblement du déficit budgétaire.

vers un modèle à l'anglo-saxonne sans le dire aux Français », en passant d'un financement par les cotisations à un financement par l'impôt. Monsieur le secrétaire d'État, dans l'expression « modèle social », il y a le mot « modèle »

Le déficit structurel, et donc l'effort structurel, reposent sur la notion de croissance potentielle, indicateur non observable consistant à apprécier ce que serait la croissance économique d'un pays si tous les facteurs de production étaient mobilisés à 100 %.

que vous soulevez mérite d'être étudiée soigneusement. En réalité, lors de leur réunion informelle en avril à Amsterdam, les ministres ECOFIN ont déjà abordé ce sujet. Ils ont invité la Commission et les États membres à réexaminer la méthodologie de calcul calcul de la croissance potentielle et de l'écart de production. [ ...] Les ministres ont convenu que les mérites d'un horizon de temps plus long sur lequel se fonder pour effectuer ces prévisions devraient être explorés dans le cadre d'une discussion technique approfondie. Cet amendement tend à recalibrer le solde structurel de 2017 sur la base des constats que je viens de rappeler. Il s'agit de s'inspirer des corrections engagées par le FMI dès 2013 pour le calcul du solde structurel. Sur la base du solde structurel recalibré pour 2017,

transparence et de démocratie. Pour 2019, le montant du prélèvement sur recettes est estimé à 21,5 milliards d'euros, contre 19,9 milliards d'euros inscrits en loi de finances pour 2018. Si l'on y ajoute 1,7 milliard d'euros de droits de douane, la contribution totale de la France s'élève à 23,2 milliards d'euros. Pour la seconde année consécutive, le montant du prélèvement européen est en hausse. Il atteint même un niveau inégalé depuis 2014. Les causes de cette hausse sont bien connues. Elles tiennent essentiellement à un effet de rattrapage de la consommation des crédits européens, en particulier de ceux dédiés à la politique de cohésion et au développement rural. Mes chers collègues, réjouissons-nous de cette augmentation, qui devrait profiter à nos territoires. À ce propos, je vous rappelle qu'en 2017 la France était, en volume, le troisième contributeur net au budget européen, mais surtout le premier bénéficiaire net en volume. Ainsi, en 2017, 13,5 milliards d'euros du budget européen ont été dépensés en France, principalement au titre de la politique agricole commune,

L'évaluation inscrite dans le projet de loi de finances est, en réalité, bien fragile. Elle dépend des prévisions de l'Union européenne, des éventuels budgets rectificatifs et des corrections apportées aux exercices antérieurs. L'année 2017 nous a montré à quel point cette évaluation était difficile à établir : l'écart entre la prévision et la réalisation a dépassé les 2,3 milliards d'euros. Il semble que nos partenaires européens se heurtent aux mêmes difficultés que nous pour évaluer le montant de leur contribution. La seconde inquiétude est suscitée par les difficultés rencontrées, ces dernières années, pour le versement des primes de la PAC aux agriculteurs et par le retard du décaissement des crédits européens pour le développement rural. Ces problèmes sont particulièrement criants pour certains programmes, comme le programme LEADER : sur 700 millions d'euros prévus pour la période 2014-2020,

le plus à en bénéficier. Ces retards contribuent à l'augmentation du « reste à liquider », qui devrait d'ailleurs atteindre le niveau record de 300 milliards d'euros en 2020, soit près de deux fois le budget annuel de l'Union européenne ; on mesure l'impact négatif de ces retards sur les dynamiques économiques des territoires qui doivent être accompagnés dans leur développement. Madame la ministre, cette situation est incompréhensible pour nos concitoyens. Il est urgent d'y remédier ! J'en viens au budget de l'Union européenne pour 2019. Lundi dernier, les négociations entre le Conseil et le Parlement européens ont échoué, de façon inattendue, en raison d'un blocage quant à l'utilisation des crédits du programme de recherche « Horizon 2020

Au-delà du budget européen pour 2019, c'est évidemment le prochain cadre financier pluriannuel qui définira l'évolution de la contribution de la France. Dans le contexte actuel de désordre mondial, marqué par une guerre commerciale qui s'aiguise, la multiplication des conflits, l'importance des flux migratoires

parfois désespérés : en témoigne, en ce moment, le mouvement des « gilets jaunes ». Le sentiment d'abandon qu'éprouvent les peuples européens se traduit, sur le plan politique, par la montée des populismes, le Brexit et la conduite, par certains États, de stratégies individuelles ou de repli sur soi. Les risques sont donc devant nous. Le cadre financier pluriannuel doit traduire des orientations politiques fortes.

À plusieurs reprises, j'ai appelé à faire preuve de plus d'ambition dans la définition du plafond de dépenses de l'Union européenne. J'espère que les élections européennes permettront d'avoir un véritable débat sur l'avenir de l'Europe. En attendant, je me réjouis que le Parlement européen se soit, de nouveau, exprimé en faveur d'un cadre financier pluriannuel s'élevant à 1,3 % du revenu brut de l'Union européenne. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que la France ne s'opposera pas à une légère augmentation de sa contribution à l'avenir ? ? La commission des finances s'est également penchée sur la question des investissements, notamment portuaires, qui devront être réalisés en France à la suite du Brexit. Ces investissements seront-ils financés uniquement par la France ? Pouvez-vous nous apporter des précisions à cet égard ? En conclusion, au-delà des observations formulées et sur la base d'une approche strictement budgétaire et comptable, je recommande, au nom de la commission des finances, l'adoption sans modification de l'article

en tant que rapporteur spécial ; il vient de nous présenter avec clarté les enjeux de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Comme l'an passé, cette contribution augmente, mais, paradoxalement, les causes de cette hausse sont vertueuses : l'utilisation des crédits européens s'accélère enfin, et les projets financés par la politique de cohésion et de développement rural prennent leur essor, cinq ans après le début de l'actuelle programmation ! Il y a quelques mois ont débuté les négociations relatives au prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, dont la Commission a dévoilé le projet en mai dernier. Ces négociations sont difficiles sens, il est illusoire d'espérer une adoption définitive avant les élections européennes de 2019. Ce projet de cadre financier pluriannuel est le fruit d'obligations et de contraintes nouvelles, qui doivent conduire à des réformes longtemps retardées. Ces obligations et ces contraintes sont connues. Il s'agit tout d'abord de la chute des recettes que va entraîner le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il s'agit ensuite des nouvelles priorités politiques qui ont émergé au cours des dernières années et auxquelles il n'a pas été possible d'apporter de réponse satisfaisante pendant l'actuelle programmation budgétaire sécurité, frontières et migrations, jeunesse, recherche et innovation. Le projet pour 2021-2027 leur accorde une large place. Malgré des recettes moindres et des priorités nouvelles, il n'est pas concevable que les politiques dites « traditionnelles », à savoir la PAC et la politique de cohésion, soient sacrifiées ou marginalisées. est la troisième obligation politique que devra respecter la prochaine programmation. La France s'est déjà battue, et doit encore se battre, pour défendre la ligne rouge que représente, pour elle comme pour beaucoup d'États partenaires, la réduction des crédits de la PAC. Devant ces contraintes, plusieurs réformes sont enfin à portée de main. En premier lieu, les nouvelles ressources propres devront faire du budget de l'Union un enjeu de « valeur ajoutée européenne » plus politique que celui du seul « juste retour

À cette unité du Parlement européen répond cependant une division cacophonique des États membres. Deuxièmement, si, comme on peut le craindre, le prochain cadre financier pluriannuel n'est pas adopté avant les élections de 2019,

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, en préambule, je voudrais rappeler combien nous regrettons la moindre place concédée, dans cette enceinte, aux débats sur la politique européenne, lesquels se dérouleront de plus après le Conseil européen des 14 et 15 décembre réduire à deux minutes les temps d'intervention en séance révèle l'intérêt porté à la question européenne dans cet hémicycle À moins de 185 jours des élections du 26 mai 2019, je prends donc la liberté de mettre à profit ces cinq minutes de temps de parole pour vous faire part de mon grand trouble : il me faut donner un avis technique et comptable sur le prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni s'apprête à quitter celle-ci et que le prochain scrutin risque d'installer au Parlement européen une majorité de députés hostiles aux valeurs humanistes qui, malgré le rejet croissant de l'Europe par les peuples, auraient pu nous mobiliser encore pour la défendre. Il nous est donc demandé de nous prononcer sur la contribution française à un budget pour lequel les conséquences de la sortie du Royaume-Uni ne sont pas connues, et dont nous ne savons pas quelle utilisation politique en fera la future majorité du Parlement européen. À ces incertitudes majeures s'ajoute le désaccord entre le Conseil et le Parlement européens, qui oblige la Commission à tenter de trouver un compromis entre deux propositions de budget

L'élaboration de ce dernier budget de la mandature du Parlement européen aurait pu être l'occasion d'une discussion sur le fond et d'une réflexion sur le projet européen. une seule priorité fait consensus : la protection des frontières extérieures et la gestion du phénomène migratoire. Pour le reste, l'action de la Commission européenne semble essentiellement concentrée sur le rejet du budget italien, dont la seule conséquence sera de renforcer le camp de ses opposants. Ces petites querelles semblent indifférentes, au regard des crises majeures que l'Europe va affronter. Elles ne sont pas dignes des espoirs placés dans la construction européenne par les générations sorties du chaos de la dernière guerre. Elles m'évoquent une oeuvre du poète grec Constantin Cavafy, dont je vous lis deux extraits : « Qu'attendons-nous, rassemblés sur l'agora ? « On dit que les Barbares seront là aujourd'hui. « Pourquoi cette léthargie, au Sénat ? « Pourquoi les sénateurs restent-ils sans légiférer ? « Parce que les Barbares seront là aujourd'hui. « À quoi bon faire des lois à présent ? « Ce sont les Barbares qui bientôt Pourquoi ce trouble, cette subite inquiétude ?-Comme les visages sont graves ! « Pourquoi places et rues si vite désertées ? « Pourquoi chacun repart-il chez lui le visage soucieux ? Parce que la nuit est tombée et que les Barbares ne sont pas venus « Et certains qui arrivent des frontières « Disent qu'il n'y a plus de Barbares. « Mais alors, qu'allons-nous devenir sans les Barbares ? « Ces gens étaient en somme une solution. Comme sur l'agora de Constantin Cavafy, il semble que l'évocation des barbares, ceux de l'intérieur pour certains, ceux de l'extérieur pour d'autres, soit devenue l'unique préoccupation d'élites incapables de proposer aux citoyennes et aux citoyens un projet transcendant qui puisse nous éviter à la fois les replis nationalistes et la gestion libérale et technocratique honnie d'une part toujours plus importante des peuples européens. Écoutez la jeunesse. Son désir d'Europe est ambitieux, généreux et prometteur. Elle s'est forgée progressivement, dans la tourmente des renoncements successifs, une conscience européenne nouvelle qui demande, pour les citoyens de cette Union future, plus de droits sociaux, plus de solidarité entre les territoires, une défense sans compromis des libertés individuelles, une association étendue et renouvelée au fonctionnement démocratique des institutions européennes et, au-dessus de tout, une action d'envergure en faveur de l'environnement et du climat : l'Union européenne est le seul espace et la seule institution dans lequel et par laquelle il serait possible d'agir efficacement pour sauver notre humanité en danger.

Cependant, notre pays étant l'un des principaux contributeurs aux recettes perçues au titre du prélèvement européen, nous devons être attentifs aux grandes orientations budgétaires proposées par la Commission- j'y reviendrai. Avec un peu plus de 21,5 milliards d'euros, la France est aujourd'hui le troisième contributeur net au budget de l'Union européenne. Rapporté au budget national, ce montant représente 5,5 % de nos dépenses publiques nettes. Le prélèvement européen constitue ainsi le quatrième budget de l'État. Pour les détracteurs de l'Europe, cela fait beaucoup. Aussi nous semble-t-il important et utile de rappeler que la France est, en volume, le premier bénéficiaire des dépenses de l'Union européenne et que, au-delà de l'approche comptable, la solidarité, en particulier au sein de la zone euro, apporte des bénéfices qui, sans être toujours quantifiables, sont bien réels.

ministre : la modernisation des politiques, afin de les rendre plus efficaces et plus justes, la création de nouvelles ressources propres- on le sait, les ressources traditionnelles s'érodent -, la fixation de conditionnalités ou encore la suppression des rabais, lesquels ne concernent pas seulement le Royaume-Uni. Le contexte est chargé et singulier, avec le retrait du Royaume-Uni, deuxième contributeur au budget de l'Union européenne. Les négociations du prochain cadre financier pluriannuel, ainsi que les élections au Parlement européen prévues en mai 2019 et l'installation d'une nouvelle Commission compliquent l'exercice. Néanmoins, nous connaissons les grandes orientations politiques qui seront mises en oeuvre dans le cadre d'un budget européen doté, pour 2019, de 166 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 149 milliards d'euros en crédits de paiement. Parmi ces recettes, la Commission a fléché trois nouvelles ressources propres un taux d'appel de 3 % sur une nouvelle assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, une part de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des droits du système européen d'échange de quotas d'émission

les travaux avancent, et je m'en réjouis, même si la chancelière Angela Merkel, à la tête d'une coalition aujourd'hui fragile, ne s'engage que très timidement.

Enfin, s'agissant des grandes politiques qui seront financées dans les prochaines années, j'évoquerai la PAC. Comme nous le savons, il s'agit de concilier les politiques traditionnelles avec les besoins croissants aux nouvelles priorités que sont notamment la gestion des migrations, la sécurité et la défense. L'équilibre est difficile à trouver et je m'inquiète de la possible baisse des crédits alloués à la PAC : nous y sommes fermement opposés Il est indispensable de promouvoir pour l'Europe une grande ambition dans le domaine agricole et alimentaire, secteur stratégique au regard non seulement de la cohésion de nos territoires, mais aussi des enjeux démographiques mondiaux et de sécurité alimentaire. Mes chers collègues, comme l'a affirmé le Président de la République dans un discours prononcé dimanche dernier devant la chambre des députés allemande, « l'Europe doit être plus forte et plus souveraine Nous ne pouvons que le souhaiter, en espérant que nous serons en mesure de répondre aux nouveaux défis sans rien sacrifier des outils qui garantissent la solidarité européenne, laquelle est le moyen de lutter contre la montée des populismes en Europe.

quand le débat européen, central pour notre vie politique, est maintenant relégué à de rares séances de questions-réponses techniques ! Oui, chers collègues, le Sénat gagnerait à se saisir de la politique européenne.

convergence ! La contribution de la France au budget de l'Union européenne s'établit à 21,515 milliards d'euros pour 2019. Elle doit être approuvée. Que le quinquennat précédent semble loin, quand, à la fin de chaque année, l'exécution partielle des engagements budgétaires européens offrait une recette importante sans fatigue de même pour les charges d'intérêts de la dette ou la réduction des dotations aux collectivités. Toutes ces économies réalisées sans grand effort et sans mérite ont été brûlées dans l'augmentation des dépenses publiques Avec une meilleure exécution en fin de mandat de la Commission, notre budget pour 2019 devra, à l'inverse, absorber une augmentation de la contribution au budget

celui de notre pays sera de 390,8 milliards d'euros, auxquels s'ajouteront plus de 500 milliards d'euros pour le budget social : c'est clairement l'inverse de ce dont notre opinion publique est probablement convaincue.

L'Europe dépend de la contribution des États plus encore que nos collectivités ne dépendent des dotations de l'État. L'autonomie fiscale revendiquée par les collectivités locales françaises est aussi un sujet

numérique. Les solutions à nos principaux problèmes sont largement européennes. La maîtrise des migrations, par exemple, ne se joue pas à l'échelle d'un seul État, mais met en oeuvre plusieurs modes d'action convergents à celle du continent européen. Les États-Unis, la Chine, la Russie, parmi d'autres pays, ont engagé un nouveau cycle historique et, à ce titre, probablement durable, dans lequel le rapport de force est devenu une forme de norme sociale mondiale.

qui ont constitué au fil du temps la première économie et le premier marché mondial et qui, instruits par les souffrances de l'histoire, connaissent l'importance d'une régulation multilatérale ou les risques engendrés par des inégalités économiques toujours plus grandes. C'est dire, mes chers collègues, que le bon

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le début de nos échanges sur le projet de loi de finances pour 2019 nous amène, tout naturellement, à examiner l'article 37 relatif à la participation de la France au budget de l'Union européenne. C'est un sujet de première importance, sachant que la France est le deuxième contributeur net européen, après l'Allemagne, avec 20,6 milliards d'euros versés en 2018. Notre participation au budget européen représente ainsi environ 15 % de l'ensemble des contributions nationales. En retour, la France a bénéficié de 14,5 milliards d'euros de dépenses, soit 11 % des dotations accordées aux États membres. par exemple- il faut le souligner -, le premier bénéficiaire des dépenses de la politique agricole commune, avec une dotation européenne de près de 9 milliards d'euros. Tout en modernisant la PAC, il est donc d'un intérêt majeur, pour nos agriculteurs et pour notre pays tout entier, que son montant soit préservé dans le futur cadre financier pluriannuel. Je voudrais ici rappeler à ceux qui fustigent la prétendue « gabegie de Bruxelles » que l'Union européenne redistribue la quasi-intégralité de ses moyens aux États membres seulement des dépenses européennes sont consacrées au fonctionnement administratif des institutions. Néanmoins, certaines critiques sont justifiées. En matière de budget européen, le n'est plus possible. Nous sentons bien que l'action quotidienne de l'Union européenne, tellement indispensable pour de nombreux projets locaux, n'est pas mesurée à sa juste valeur par les Français. Il faut que les dépenses de l'Union européenne soient plus visibles, plus proches des citoyens, davantage tournées vers leurs préoccupations concrètes. Il est plus que temps de donner à l'Union européenne les moyens d'agir. Le rapport Monti de l'année dernière a tiré la sonnette d'alarme quant à l'urgence de réformer le budget européen. Le Parlement européen a pris récemment des positions très fortes sur le futur cadre financier pluriannuel, en réclamant un budget s'établissant à 1,3 % du RNB des États membres, ce qui serait du jamais-vu.

Dans l'idéal, le prélèvement sur recettes que nous examinons aujourd'hui ne devrait plus exister, ou en tout cas ne constituer qu'une part marginale du financement de l'Union Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais je ne retiendrai que les plus réalistes à court terme : attribuer à l'Union européenne une part de l'assiette harmonisée de l'impôt sur les sociétés, les recettes tirées du système européen d'échanges de quotas d'émission, une taxe sur les bénéfices des GAFA ... Après le Brexit, il faudra également mettre fin à la logique des rabais sur les rabais, qui grève le budget de l'Union. Concernant les dépenses, le budget de l'Union européenne doit mieux prendre en compte les priorités des Européens et être tourné vers l'avenir. Une des priorités doit être d'assurer la protection des Européens, en consacrant plus de moyens à la gestion des frontières de l'Union et à la défense européenne. Le budget européen doit également contribuer à faire de notre économie une économie de la connaissance performante et compétitive. cette fin, nous soutenons une hausse des crédits destinés à l'innovation, à la recherche et au marché unique du numérique. Soyons réalistes : face aux géants américains ou chinois, seule une stratégie européenne commune en matière d'innovation nous permettra de rester compétitifs au plan mondial.

Vous avez mené des consultations auprès de nos concitoyens, qui disent peu ou prou la même chose : c'est ensemble que nous serons plus en sécurité, plus prospères et plus forts. Dans cette perspective, la France et ses partenaires doivent enfin donner à l'Union européenne les moyens de ses ambitions, qui sont immenses, à la mesure des attentes de nos concitoyens.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, heu-reux ! Heureux je suis, comme Fernand Raynaud dans son sketch éponyme, l'un des plus célèbres de sa grande carrière Je suis heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, à la tribune du Sénat, sur l'article 37 de ce PLF pour 2019 concernant le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne.

Il faut bien le dire, les occasions de ce genre sont devenues de plus en plus rares dans cette enceinte depuis que la majorité du Sénat a choisi de supprimer purement et simplement le temps d'expression politique des groupes à l'occasion des débats en séance publique qui se tenaient autrefois en amont de chaque Conseil européen. pourtant une formidable occasion à la représentation nationale, dans toute sa diversité, d'exprimer publiquement ses attentes et ses exigences envers le Gouvernement quant aux discussions européennes à venir.

passionnant pour ceux qui n'en auront pas encore lu les conclusions dans la presse ... Dans les circonstances présentes, ce souci de parcimonie du temps de parole de nos très hautes autorités sénatoriales tombe particulièrement mal ! Ce dimanche 25 novembre se tiendra en effet un Conseil européen extraordinaire consacré à la question, cruciale, de l'accord trouvé sur les conditions de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est ballot, mais notre belle et haute assemblée n'aura pas l'heur de s'exprimer publiquement, dans la diversité de sa composition politique, sur ce sujet pourtant capital. Ce qui est encore plus ballot, c'est que nous sommes à six mois des prochaines élections européennes, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles seront déterminantes pour le devenir de l'Union européenne ... Vous me connaissez, comme je suis bienveillant par nature et bienséant par devoir, je n'ose voir dans cette décision à contretemps une quelconque manoeuvre politique d'une majorité sénatoriale peut-être encore un peu agacée de n'avoir pu devenir majorité politique lors des élections de l'an aura tout de même bien une expression publique du Sénat à rebours sur ces questions européennes, puisque les séries de questions posées au Gouvernement seront introduites- en toute impartialité, cela va de soi -par des interventions de huit minutes chacune de deux ou trois présidents de commission, cela devant un hémicycle sans doute plein à craquer un lundi en début d'après-midi ... Tout cela sera très économe en temps et, n'en doutons pas, parfaitement proportionné, au regard des équilibres politiques au sein de notre assemblée. Le débat démocratique et pluraliste sur l'Europe dans cette maison en sortira très certainement grandi ! Le Sénat, qui a toujours veillé à se différencier- en bien -de l'Assemblée nationale et qui s'est longtemps enorgueilli d'organiser systématiquement de tels débats préalables à la tenue de chaque

ils sont largement détaillés dans l'excellent rapport de notre collègue Patrice Joly. Je constate avec satisfaction la montée en charge de nombreuses politiques sectorielles, notamment celles en direction de la jeunesse, avec Erasmus +, mais aussi l'augmentation de l'investissement dans l'innovation ou dans la protection des citoyens européens, avec un accent particulier mis sur la protection de nos frontières extérieures, la sécurité et l'accueil des demandeurs d'asile.

juge, à juste titre, que les grandes orientations du projet de cadre financier présenté par la Commission européenne sont, de manière générale, très en retrait par rapport aux enjeux actuels. Si des efforts vont être consentis, ce dont je me félicite, dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure, d'autres politiques, notamment en faveur de la jeunesse, comme Erasmus + ou l'initiative pour l'emploi des jeunes, des jeunes, ou dans les domaines de la recherche ou de la lutte contre le changement climatique, devraient faire l'objet de beaucoup plus de soutien. Le fait que certains pays demandent une diminution du budget européen complique bien entendu l'équation.

pour accompagner les petites et moyennes exploitations agricoles, surtout en zones de montagne et de moyenne montagne et, bien entendu, sur le pourtour méditerranéen. De même, un affaiblissement des fonds structurels serait un bien mauvais calcul. Sans ceux-ci, en effet, de nombreuses régions européennes verraient leur développement stoppé net. Un ciblage des territoires les plus fragiles permettrait, de ce point de vue, d'atteindre une plus grande efficacité, le produit intérieur brut d'un pays ou d'une grande région ne signifiant rien : en Occitanie, ma région, on sait que les Cévennes n'ont pas les mêmes besoins que le bassin toulousain, par exemple.

L'heure est venue d'agir. Nous connaissons toutes et tous les forces et les faiblesses de l'Union européenne ; il faut désormais nous mobiliser pour en faire un espace inclusif de paix, de croissance,

dépense obligatoire de solidarité entre États membres, qui représente le cinquième poste de notre budget, après l'enseignement scolaire, la défense,

intelligente et inclusive, d'une part, croissance durable et ressources naturelles, d'autre part. Viennent ensuite d'autres rubriques, telles que la sécurité et la citoyenneté, l'Europe dans le monde et l'administration, notamment. Fixer ce prélèvement constitue un exercice difficile, reconnaissons-le. La politique agricole commune et la politique de cohésion représentent toujours, respectivement, 38 % et 31 % des crédits de paiement.

10 octobre dernier, intitulé « La chaîne de paiement des aides agricoles (2014-2017) : une gestion défaillante, une réforme à mener »,

prochaine à 21,5 milliards d'euros. La France contribuera ainsi à hauteur d'environ 15 % au budget de l'Union européenne. Il faut nous rappeler que le budget européen n'est pas qu'un exercice

La politique agricole commune est particulièrement visée par une réduction de son financement dans le cadre de la programmation financière pour 2021-2027. Je me dois de rappeler que la PAC est le budget fondateur de l'Union européenne. Cette ressource est essentielle, vitale pour nos agriculteurs, qui ont aujourd'hui de plus en plus de mal à faire face à l'ensemble des charges qui pèsent sur eux. La France doit se battre pour le budget de la PAC ; il y va de la survie de nos agriculteurs

la ratification de celui-ci par le Parlement européen et le Parlement britannique. Cette semaine sera décisive, avant le Conseil européen exceptionnel de dimanche prochain, qui pourrait déboucher sur un accord définitif. Le Brexit pourrait servir de catalyseur pour réformer l'Europe et lui donner un nouveau souffle. Le peuple souhaite plus de transparence et comprendre à quoi sert l'Europe. En dehors des défis économiques et politiques, l'Europe doit relever le défi migratoire. La question migratoire est aujourd'hui à l'origine d'une profonde crise politique et humaine. La rhétorique sur la fermeture des frontières et le traitement des demandes d'asile en dehors du territoire européen est particulièrement inquiétante, à la fois pour la solidarité européenne et pour le respect de nos valeurs. L'immigration irrégulière aux frontières de l'Europe est en constante augmentation depuis 2015. L'augmentation budgétaire

je vous remercie pour ce débat, qui est un moment démocratique important permettant d'illustrer de façon concrète la valeur ajoutée des politiques européennes. Je me garderai bien, monsieur le sénateur Gattolin, d'intervenir dans un débat qui concerne une décision souveraine de la Haute Assemblée. Je confirme néanmoins l'intérêt qu'il y a, pour la France, à pouvoir s'appuyer sur la position des groupes représentés dans les deux assemblées avant de participer au Conseil européen. Il ne me sera naturellement pas possible, dans le temps qui m'est imparti, de répondre à l'ensemble des observations des différents orateurs, mais je tiens à revenir sur certaines

La même situation s'était produite voilà quatre ans pour le budget de 2015. Durant cette discussion, le Conseil a veillé à garantir le financement des priorités politiques, tout en assurant une budgétisation prudente en crédits, afin de conserver la marge nécessaire pour faire face aux imprévus en cours d'année. La négociation a échoué en grande partie en raison d'un point de principe sur la technique budgétaire, auquel le Parlement est attaché

Conformément aux stipulations du traité et comme elle l'avait fait en 2014, la Commission européenne va proposer un projet de budget révisé d'ici à quelques jours, afin qu'un budget puisse être adopté avant la fin de l'année.

Ce budget permet de préparer le prochain cadre financier pluriannuel, dont nous reparlerons, en faisant un effort sur des dépenses nouvelles. J'ajoute immédiatement que, sur les 165,6 milliards d'euros de crédits d'engagement et les 148,7 milliards d'euros de crédits de paiement du projet de budget initial, les priorités classiques que sont la PAC et la politique de cohésion restent bien évidemment les principales masses budgétaires ; nous y avons veillé attentivement.

de budget prévoit de faire monter en puissance la croissance et l'innovation, ainsi que les mesures en faveur de la jeunesse. Je pense à la montée en charge d'Erasmus +, dont M. le sénateur Sutour de permettre à de plus en plus d'étudiants, mais aussi, désormais, d'apprentis, de se former en Europe. Dans le même temps, ce budget contribuera à une meilleure politique migratoire et à un meilleur contrôle des frontières de l'Union ainsi qu'à une plus forte solidarité au-delà de celles-ci, notamment en continuant à financer l'accompagnement, l'éducation et l'hébergement des personnes qui fuient les conflits, en Syrie et ailleurs. autre priorité nouvelle et importante. L'année 2019 marquera une avancée majeure pour le volet industriel et capacitaire de l'Europe de la défense, composante incontournable de l'autonomie stratégique européenne. un programme européen spécifique permettra aux entreprises européennes d'unir leurs forces pour financer des projets en commun. Ce programme préfigure le futur fonds européen de défense, que la Commission européenne propose de doter de 13 milliards d'euros dans le cadre financier pluriannuel pluriannuel 2021-2027. Cela m'amène tout naturellement à évoquer les perspectives financières pour l'après 2020.

Je doute que nous parvenions à un accord, comme le souhaiterait la Commission européenne, avant les élections européennes ou que nous arrivions à dégager dès décembre le premier niveau de financement du prochain cadre financier pluriannuel. Ce serait d'ailleurs un étrange message que de dire aux électeurs que les priorités et les moyens budgétaires correspondants sont définis avant qu'ils se soient exprimés je l'ai rappelé le 12 novembre dernier lors du conseil Affaires générales. Le Conseil européen y reviendra au mois de décembre. Au titre des défis auxquels l'Europe est confrontée, de nouvelles priorités sont apparues ou montent en puissance

Nous sommes parvenus à mobiliser largement, et ce sont aujourd'hui vingt et un États membres qui demandent le maintien du budget de la PAC à son niveau actuel pour l'Union européenne à Par ailleurs, le budget doit traduire la solidarité de l'Union européenne et refléter ses valeurs. C'est pourquoi la France soutient, au côté de nombreux États membres, la proposition de la Commission européenne de renforcer le lien entre l'octroi de financements européens et le respect des valeurs fondamentales de l'Union Nous estimons d'ailleurs qu'il convient d'aller plus loin, afin que le budget européen puisse également favoriser la convergence des États en matières fiscale et sociale, une convergence essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. J'ajoute que nous souhaitons intégrer au cadre financier pluriannuel à vingt-sept un budget pour les dix-neuf États de la zone euro. Bruno Le Maire et son collègue allemand, Olaf Scholz, ont présenté nos idées à cet égard le 19 novembre Le départ du Royaume-Uni représente une occasion historique de remettre à plat le système de financement du budget européen. La Commission européenne a fait des propositions qui vont dans le bon sens,

une modernisation des politiques, des conditionnalités dans l'emploi des fonds, la mobilisation de nouvelles ressources propres et la suppression complète des rabais.

Ce budget est fondé sur une hypothèse : la conclusion d'un accord de retrait. Nous y sommes au niveau technique. Il est vraisemblable qu'un sommet se tiendra dimanche

signalé, une incertitude demeure sur la ratification de l'accord par le Parlement britannique. Cette incertitude est forte ; ce n'est pas la première s'agissant du Brexit, mais nous devons être prêts pour tous les scénarios.

d'ailleurs, la date à laquelle ces contrôles devront être mis en place- dès le 30 mars en cas d'absence d'accord de retrait ou à la fin de la période de transition, si la relation future justifie ces contrôles.

les investissements à réaliser, les recrutements à mener et l'organisation des futurs contrôles, dont nous avions perdu l'habitude dans le trafic transmanche. Pour ne parler que du volet européen qui nous concerne aujourd'hui, je vous confirme que nous travaillons pour que les programmes européens permettent de financer des adaptations au Brexit dès maintenant, puis, le cas échéant, dans les premières années du prochain cadre financier pluriannuel. la Commission européenne lancera le mois prochain un appel d'offres pour le mécanisme d'interconnexion en Europe, doté de 65 millions d'euros, afin de cofinancer des projets de liaisons transfrontalières et d'assurer la connexion et le développement des ports maritimes du réseau global. Nous nous mobilisons pour que le plus grand nombre possible de ports français puissent participer aux futurs appels d'offres du corridor mer du Nord-Méditerranée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Union européenne n'est pas figée, bien au contraire. Nous sommes convaincus, avec le Président de la République, qu'elle doit changer en profondeur.

déterminera au travers du prochain cadre financier pluriannuel ses grands choix politiques pour la période à venir. D'ici là, le budget européen pour 2019 donnera à l'Union européenne et à la France les moyens d'être plus efficaces, plus fortes, plus protectrices. C'est pourquoi, au nom du Gouvernement,